Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour de demain, samedi 24 juillet, le soir, de la suite de l'examen du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la crise sanitaire

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux d'engager devant la Haute Assemblée l'examen d'un projet de loi crucial dans le combat que nous menons contre cette pandémie. Je vous remercie très sincèrement

fois que je me suis présenté devant vous, nous nous trouvions dans une tout autre situation sanitaire. Nous étions alors confrontés à un variant alpha, qui nous était venu de Grande-Bretagne, nous connaissions également le variant brésilien, un variant sud-africain et nous étions loin d'imaginer qu'un variant venu d'Inde, appelé delta, allait progressivement, mais très rapidement, se répandre sur toute la planète.

des études publiées cette semaine attestent une charge virale mille fois plus élevée, ce qui est extrêmement important, dans la mesure où la charge virale est un des reflets de la contagiosité.

ils fréquentent peut-être un peu plus les milieux festifs, ils ont beaucoup de relations sociales et ils ne sont pas suffisamment vaccinés. L'été dernier, nous avions constaté la même situation, mais dans des proportions bien moindres. Souvenez-vous, l'épidémie était repartie par la jeunesse et avait ensuite touché les catégories les plus âgées, entraînant une deuxième vague.

Néanmoins, cela laisse encore 12 millions de personnes vaccinables qui ne le sont pas. Surtout, parmi les populations fragiles, âgées et/ou atteintes

semaines. Jusqu'ici, nous connaissions deux scénarios. Le premier est le confinement : nous fermons l'accès à tous les espaces culturels, sportifs, économiques pour tous les Français. C'est la distanciation sociale poussée à son paroxysme, de sorte que les gens ne se contaminent plus. L'épidémie reflue et nous avons vaincu la vague. La deuxième option, et certains pays ont fait ce choix, est de considérer que, au vu du taux de couverture vaccinale et dans la mesure où la vaccination a été proposée à un grand nombre de Français,

sans se poser trop de questions et en croisant les doigts ne me semble pas être un choix conforme à la philosophie de notre pays et de notre protection sociale.

Telle est la logique du dispositif. Nous souhaitons pouvoir l'appliquer le plus tôt possible, de manière à limiter les risques d'explosion de la vague épidémique et à éviter les situations d'urgence qui pourraient nous contraindre à mettre en place des mesures pouvant aller jusqu'à des fermetures administratives. Vous avez sans doute constaté que, dans certains départements, notamment les Pyrénées-Orientales, ont déjà été décidées des fermetures d'établissements recevant du public, à partir de vingt-trois heures. Nous ne souhaitons pas diffuser ces mesures dans les autres départements touchés, mais en rester à la gestion par le passe sanitaire.

Cette population professionnelle très large connaît un taux de couverture vaccinale variable : chez les médecins et les pharmaciens, on atteint plus de 90 % de vaccinations complètes,

sont moins vaccinées que la population générale. Même si l'on utilise le masque, même si l'on fait très attention parce que l'on ne veut contaminer personne, même si l'on se lave les mains très régulièrement ou que l'on utilise du gel hydroalcoolique, le risque de faire entrer le virus dans un établissement pour personnes âgées ou dans un hôpital

sur un clivage politique, puisque chaque gouvernement, en responsabilité, en son temps, a été amené à prendre cette décision difficile, mais nécessaire. J'ai réuni les sept ordres professionnels les huit fédérations d'établissements de santé, qui se sont engagés par écrit, en considérant que la vaccination, lorsque l'on soigne et que l'on prend soin des personnes fragiles, relevait d'une obligation morale, éthique, professionnelle et déontologique, et que l'on pouvait, s'il le fallait, la rendre obligatoire.

40 %. C'est un problème, parce que si vous sortez chez vous alors que vous êtes contagieux, l'épidémie ne va pas s'arrêter, c'est une certitude ! C'est pourquoi nous vous proposons une disposition qui va plus loin que ce que nous avons fait jusqu'à présent et qui se rapproche des décisions prises dans d'autres pays

plus ou moins positivement, mais toujours de manière constructive, les transformations profondes apportées en commission sénatoriale, dans l'attente de pouvoir en débattre avec vous. J'oublie un dernier point : vous avez supprimé le recours au passe sanitaire dans les grands centres commerciaux,

Madame le président, madame, monsieur les ministres, madame, monsieur les présidents de commission, madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues, la flambée de l'épidémie justifie la mise en oeuvre de mesures d'urgence et d'exception pour lui donner un coup d'arrêt. Avec déjà plus de 20 000 contaminations journalières, la vague est de grande ampleur

Faut-il réellement attendre la preuve par neuf, c'est-à-dire une forte augmentation du nombre de victimes, pour agir ? C'est un risque que je ne vous proposerai pas de prendre. Faut-il alors confiner la France une quatrième fois ? Chacun d'entre nous voudrait l'éviter. Le Gouvernement nous propose de tenter de le faire par la combinaison de trois moyens : l'obligation du passe sanitaire pour l'accès à certains lieux, la mise à l'isolement forcé de nos concitoyens contaminés, la vaccination des professionnels au contact de personnes vulnérables. Nul ne peut dire que cela sera suffisant, mais je vais vous recommander de donner ses chances à ce dispositif en vous proposant, toutefois, de le rendre plus simple, plus clair, plus efficace plus respectueux des libertés. Je vais donc vous proposer de prendre position sur six questions essentielles. La première est celle du cadre de l'action des pouvoirs publics. Sommes-nous toujours dans la gestion de la sortie de l'urgence sanitaire ou sommes-nous revenus dans l'état d'urgence sanitaire lui-même ? Il est clair qu'un régime de pouvoirs exceptionnels justifié par une flambée

ne peut être mis en place légitimement que par le retour à l'état d'urgence sanitaire. La privation de droits fondamentaux pour toutes les personnes qui ne peuvent produire un passe sanitaire, l'obligation vaccinale imposée à des catégories très larges de professionnels, la mise à l'isolement des porteurs du virus constituent des mesures tellement exorbitantes du droit commun, en démocratie, que celles-ci ne sont concevables qu'à titre temporaire, dans le cadre d'une urgence sanitaire reconnue et sous un contrôle parlementaire et juridictionnel accru. La deuxième question est celle de la durée de l'habilitation donnée par le Parlement pour l'application de ces mesures. le Gouvernement, monsieur le ministre, à maintenir de sa propre initiative, et à sa discrétion, pendant une durée de plus de cinq mois, un régime d'exception frappant massivement les Français dans leurs droits essentiels. Cela créerait un précédent dangereux pour le traitement des crises de toute nature auxquelles notre Nation ne manquera pas d'être confrontée à l'avenir.

mes chers collègues, de ne consentir les pouvoirs exceptionnels demandés par le Gouvernement que jusqu'au 31 octobre prochain et non jusqu'au 31 décembre. Au 31 octobre, de deux choses l'une : soit le pari risqué d'une maîtrise de l'épidémie aura fort heureusement été gagné et il ne sera pas utile de maintenir, à un tel degré, la suspension de libertés jusqu'au 31 décembre ; soit, au contraire, l'épidémie n'aura pas été jugulée et des mesures supplémentaires devront être prises- ou l'auront d'ailleurs déjà été -, et ce sera si grave que que cela ne pourra être fait sans une nouvelle autorisation du Parlement. Dans les deux cas, c'est au Parlement de décider sans déléguer son pouvoir. Le corollaire, et c'est la troisième question que je vous demanderai de trancher, c'est que, compte tenu de la gravité de la situation, si le Gouvernement décidait- il ne le souhaite pas, et nous non plus -de rétablir le couvre-feu ou le confinement sur tout ou partie du territoire national- et il le peut déjà ! -, il faudrait que le décret qu'il prendra ne puisse s'appliquer au-delà d'un mois sans autorisation du Parlement. Pour exercer notre contrôle, nous devrons aussi demander au Gouvernement d'évaluer et de rendre publics chaque semaine les résultats de l'action que nous l'autoriserons à mettre en oeuvre. Nous pourrons alors, s'il y a lieu, délibérer de manière éclairée pour déterminer s'il faut une nouvelle loi. Quatrième question : comment contrôler et sanctionner l'obligation de présentation du passe sanitaire ? Le Gouvernement nous propose un dispositif reposant sur des sanctions pénales. Celles-ci étaient à l'origine tout à fait disproportionnées. Le Conseil d'État y a mis bon ordre, mais c'est le dispositif lui-même qui me paraît devoir être revu pour plus d'efficacité. Au lieu de prévoir un régime pénal, qui risque de ne pas être efficace en raison de sa lenteur et des incertitudes sur le prononcé des sanctions, je vous propose un régime de police administrative très simple : mise en demeure de se conformer aux obligations prévues par la loi sous

Le système sera rapide, dissuasif et donc efficace. Cinquième question : comment assurer l'effectivité de l'isolement des personnes contaminées au lieu d'hébergement de leur choix ? Là encore, le Gouvernement me semble inutilement répressif, comme si la peur du gendarme et du juge était susceptible de régler tous les problèmes. Il veut aussi que la police et la gendarmerie aient accès, les préfectures, au fichier de santé publique dont nous avons autorisé la création l'an dernier pour l'identification et la protection des personnes qui ont été exposées à une contamination, et ce afin de contrôler l'isolement des personnes contaminées et de faire sanctionner sa violation.

Je vais donc vous proposer une autre répartition des tâches. D'ailleurs, vous l'avez vous-même esquissée, monsieur le ministre : les agents de l'assurance maladie qui gèrent les plateformes chargées du traçage et ceux qui gèrent le contrôle des arrêts de travail pour maladie procéderont à des contrôles téléphoniques et sur place. S'ils constatent ou soupçonnent que l'isolement n'est pas respecté, ils saisiront l'agence régionale de santé pour qu'un arrêté préfectoral de placement à l'isolement soit immédiatement pris. Cet arrêté sera notifié à la police ou à la gendarmerie du lieu d'hébergement. Alors et alors seulement, c'est-à-dire par exception, une procédure répressive pourra effectivement être mise en oeuvre sans que jamais les préfectures aient eu accès au fichier des personnes contaminées. Sixième question : faut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous les adultes ? Cette hypothèse est parfois présentée comme une alternative au dispositif proposé par le Gouvernement. Ce n'est pas le cas de mon point de vue. L'obligation vaccinale ne peut en effet donner un coup d'arrêt, ici et maintenant, à la flambée actuelle de l'épidémie. Obligation ou pas obligation, il faut plusieurs mois pour immuniser les millions de Français qui ne le sont pas encore. Pendant ce temps, l'épidémie exploserait. Qui plus est, il ne suffit pas de déclarer la vaccination obligatoire pour qu'elle soit effective. Ce n'est pas la même chose le ministre a justement mis en évidence l'impossibilité matérielle de la contrainte, si elle doit s'exercer sur des millions d'individus en même temps. L'obligation risquerait donc de n'être que proclamatoire. Rien n'interdirait d'approfondir ce débat dans les mois qui viennent, si des solutions étaient trouvées pour surmonter ces obstacles. Pour le moment, l'essentiel est de réenclencher une dynamique de vaccination massive,

et leur autonomie de décision, de ne pas les infantiliser ni les traiter comme des délinquants en puissance. L'État est d'abord là pour entraîner et convaincre, pas pour punir, sanctionner et contraindre. La réussite

n'aurons jamais assez de policiers, de gendarmes et de juges pour contrôler et sanctionner la masse immense des situations où les mesures sanitaires seront appliquées. À la fin, c'est donc bien la libre volonté des Français qui sera déterminante.

mes chers collègues, la France fait face, depuis le début du mois de juillet, au risque d'une nouvelle vague épidémique d'une ampleur potentiellement inédite. Ce risque coïncide avec la diffusion rapide du variant delta, sensiblement plus transmissible que les précédents variants, ainsi qu'avec un ralentissement du rythme de la vaccination au mois de juin dernier. Dans ce contexte, je partage les deux constats posés par le Gouvernement dans son projet d'une part, une réaction urgente s'impose pour freiner cette reprise ; d'autre part, la vaccination est notre meilleure arme pour lutter contre l'épidémie. Ne nous leurrons pas : l'extension du passe sanitaire constitue une incitation particulièrement puissante à la vaccination en population générale. Certains y verront même une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom. Peu importe comment on la qualifie, la commission soutient sans complexe cette stratégie, qui lui apparaît pleinement justifiée au regard de la reprise épidémique brutale, alimentée par le variant delta.

Au-delà de l'obligation vaccinale des professionnels en contact avec des personnes vulnérables, il appartient donc à l'ensemble des pouvoirs publics de faire oeuvre de pédagogie et d'exemplarité pour emporter l'adhésion massive de la population au seul outil qui nous permettra de sortir durablement de cette crise. Dans cet exercice que je sais délicat, monsieur le ministre, vous pouvez compter sur le soutien déterminé de très nombreux parlementaires, qui sont prêts à porter le message suivant : les vaccins contre la covid-19 sont très efficaces et sûrs. J'en viens aux modifications apportées par la commission des affaires sociales. L'article 5 prévoit la vaccination obligatoire des catégories de professionnels ou de personnel en contact avec des personnes vulnérables. La commission des affaires sociales souscrit à l'idée selon laquelle cette obligation vaccinale contre la covid-19 participe du devoir d'exemplarité, mais aussi du devoir éthique qu'ont les soignants de ne pas nuire et de protéger les personnes vulnérables qu'ils sont amenés à prendre en charge.

En revanche, elle a veillé à garantir que l'expertise de la Haute Autorité de santé soit mobilisée sur la détermination des justificatifs attestant la satisfaction de l'obligation vaccinale, ainsi que sur une éventuelle décision par laquelle le Gouvernement serait conduit à suspendre cette obligation. L'article L'article 6 définit les conditions de présentation de la satisfaction à l'obligation vaccinale pour les personnes concernées. À cet égard, la commission a renforcé la protection du secret médical et sécurisé les modalités de transmission et de conservation des informations tirées du contrôle des justificatifs. À l'article 7, la commission a étendu les souplesses destinées à permettre aux professionnels soumis à l'obligation vaccinale de poursuivre leur activité en se conformant à cette exigence dans des délais raisonnables. Elle a ainsi prévu une période complémentaire du 15 septembre au 15 octobre 2021, pendant laquelle les professionnels pourront continuer à travailler, même si leur vaccination n'est pas complète, dès lors qu'ils auront démontré leur volonté de se faire vacciner, par l'administration d'une première dose, et sous réserve, bien entendu, de présenter le résultat négatif d'un test virologique. Il convient en effet de ne pas faire de la date du 15 septembre un couperet punitif et de tenir compte des difficultés que pourraient rencontrer les professionnels pour se faire vacciner dans les délais. Par ailleurs, la commission a précisé les conséquences pour l'emploi qui devront être tirées de l'interdiction d'exercer pour défaut de vaccination. La suspension des fonctions ou du contrat de travail, assortie d'une interruption du versement de la rémunération, constitue en effet la sanction la plus équilibrée. Elle est une incitation puissante à ce que les professionnels les plus réticents rejoignent les rangs de leurs collègues vaccinés. En revanche, un licenciement à l'issue de deux mois de suspension paraît manifestement disproportionné. C'est pourquoi la commission est revenue sur la création d'un motif spécifique de licenciement, tiré de la persistance du refus de se faire vacciner, au-delà d'une période d'interdiction d'exercer de deux mois. Enfin, l'article 9 prévoit une autorisation d'absence pour un salarié ou un agent public qui se rend à un rendez-vous de vaccination contre la covid-19. La commission a étendu cette autorisation d'absence aux salariés et agents publics qui doivent accompagner leurs enfants éligibles à la vaccination. Tel est

Madame le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce passe ou plutôt cet sanitaire que l'on nous demande de voter est le parfait symbole du quinquennat, un quinquennat qui aura été jalonné par les injures et le mépris de l'exécutif envers le peuple français ! Souvenons-nous réfractaires », « fainéants », « mafieux », « gens qui ne sont rien », « illettrés », « alcooliques », encore récemment « capricieux » et « défaitistes », et j'en oublie sûrement ... Quand le pays réel a dit stop, quand il est descendu sur les ronds-points vêtu de ce gilet jaune de détresse, l'Élysée a répondu par la plus violente répression qu'un mouvement social ait eue à subir depuis des décennies. Le peuple français, ne vous en déplaise, monsieur le ministre, est enraciné : il est attaché à son pays, à son histoire, à son identité, à sa liberté. Incapable de comprendre les Français, le Gouvernement a aussi été incapable de le convaincre de l'efficacité de sa politique sanitaire. Il est vrai qu'il a multiplié les fiascos : investissements dans l'hôpital public sacrifiés, mensonges et échecs lamentables sur les masques- rappelez-vous qu'il suffisait d'éternuer dans son coude pour éviter la contamination ! -, refus dogmatique de fermer les frontières, incapacité à mettre des tests à la disposition de nos concitoyens, changements d'avis permanents ... Le Gouvernement s'est donc rabattu sur la seule arme qui lui restait : l'enfermement généralisé, le confinement. Et pendant que la racaille ethnique continue de faire régner le chaos et la terreur, que les islamistes conquièrent chaque jour de nouveaux territoires, le Gouvernement reste impitoyable ... mais avec les honnêtes gens. Aujourd'hui, il veut à nouveau faire usage de la trique et diffuse plus encore le virus mortel de la division de la Nation, en prévoyant une obligation de vaccination, qui ne dit pas son nom, et la mise en place d'une société de surveillance généralisée où chacun, vacciné ou non, devra sortir son passeport sanitaire dix fois par jour pour aller acheter son pain ou, tout simplement, voir sa famille. Quant aux non-vaccinés, qui ont le droit de ne pas l'être- j'y insiste -, ils deviendront de fait des citoyens de seconde zone, assignés à résidence. Ils sont d'ailleurs déjà considérés comme des délinquants. Alors non,

Alors que les pompiers, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes comptent leurs morts pour avoir été en première ligne depuis le début de cette guerre contre la pandémie, alors qu'ils ont manqué de tout tout par votre faute, vous commettez l'infamie de les culpabiliser et de les diffamer, allant même jusqu'à les menacer de les licencier s'ils ne se soumettent pas à votre diktat sanitaire. Mais c'est de la folie ! c'est de la folie ! C'est inacceptable ! Honte à ce gouvernement de menteurs, de diviseurs, de manipulateurs, qui tente de faire oublier que le seul responsable de cette catastrophe sanitaire, c'est lui

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, en écoutant notre collègue Ravier, j'ai soudain compris que nous vivions sous le joug d'une dictature et que, sans une poignée d'héroïques résistants, nous ne nous en serions pas aperçus. On nous a tous inoculé dès notre plus jeune âge le DT Polio. Depuis, Agnès Buzyn, cette autocrate, a imposé huit vaccins obligatoires. Le carnet de vaccination, ancêtre du passe sanitaire, instaurait un contrôle généralisé de la population. population. avait décidé qu'aucun enfant- tenez-vous bien ! -ne pouvait entrer à l'école sans cet, pour parler comme M. Ravier. Notre droit le plus sacré à choisir la maladie plutôt que l'immunité était bafoué depuis Pasteur. Les Français eux-mêmes avaient intériorisé la servitude, pensant, comme Hobbes, que seul un Léviathan armé de seringues et d'aiguilles pouvait les sauver. Heureusement, comme Zorro, Facebook et Twitter sont arrivés, permettant à une avant-garde éclairée de se regrouper contre le totalitarisme vaccinal. Après que, durant des années, onze vaccins nous ont été injectés à l'insu de notre plein gré, au douzième, bingo ! Nos yeux se sont dessillés grâce à ces combattants de la liberté qui ont eu le courage de nommer l'infamie du passe sanitaire

En définitive, la meilleure preuve des progrès de l'humanité, c'est qu'en 2 500 ans nous sommes passés de Socrate sur l'agora à Francis Lalanne sur Facebook. Quel dommage que les réseaux sociaux n'aient pas existé plus tôt pour défendre contre les dictateurs de la piqûre la liberté de mourir en harmonie avec la nature et ses dons, parmi lesquels nos compagnons de toujours, la variole, la poliomyélite, la peste et le choléra, qui ont permis aux plus grands auteurs, Camus, Giono, Thomas Mann et d'autres d'écrire les chefs-d'oeuvre immortels de la littérature de pandémie La variole a disparu ; la covid-19, elle, a des chances de survivre grâce à tous les résistants numériques, qui exigent le droit d'attraper le virus et de le combattre, comme les Polonais de 1940 contre les chars soviétiques, à la seule force de leurs poitrines et de leurs mains nues, et avec le seul secours de l'hydroxychloroquine, parfois renforcée par un médicament redécouvert, le Ricard ! Les anciens mouraient le poing levé sur les barricades en chantant ; nos héros sont prêts à mourir le poing levé dans les discothèques au son de ... Comment Comment ne pas admirer aussi cette députée, qui a fait le choix cornélien de fausser compagnie à la majorité sans laquelle elle n'aurait jamais été élue et de haranguer, nouvelle Liberté guidant le peuple, les foules de résistants à la dictature sanitaire en les invitant, comme Henri IV, à se rallier à son panache blond et à envahir les permanences de ses collègues favorables au passe sanitaire. Je voudrais, cette fois plus sérieusement, implorer que l'on veuille bien nous épargner cette mauvaise querelle sur les libertés. Ce n'est pas le Gouvernement, le pouvoir médical ou les partisans de la vaccination obligatoire qui les restreignent, c'est la pandémie. Loin d'être un viol de notre liberté, les mesures annoncées sont les conditions de son rétablissement. Vaccination accélérée ou confinement dans deux mois, telle est l'alternative, comme l'a très bien compris la grande majorité des Français qui réalisent que c'est en limitant quelques libertés aujourd'hui que l'on a une chance d'en sauver de bien plus précieuses en septembre C'est donc ce que nous allons faire, et ce choix ne fait pas du Président de la République un dictateur, mais un décideur. Il ne fait pas du Parlement un rassemblement de tyrans, mais une assemblée de responsables. Cette décision est-elle difficile ? Elle est au contraire limpide. Le vaccin est une prouesse scientifique que des milliards d'êtres humains attendent désespérément. Quel gouvernement serait assez irresponsable pour ne pas le proposer à tous, le plus vite possible, et pour ne pas protéger en attendant ceux qui ne le sont pas encore ? Il ne reste donc que des questions de méthode, ce qui ne les rend pas plus simples pour autant.

ne pourra être menée à son terme avant plusieurs mois, alors que le temps presse- Philippe Bas a raison. L'épidémie flambe de manière exponentielle. Les Chinois viennent de découvrir que la charge virale du variant delta est mille fois supérieure à celle des précédents variants. Et nous serons dans quelques jours à 40 000 ou 50 000 cas quotidiens. Le Gouvernement a choisi le passe sanitaire, estimant que celui-ci serait mieux accepté. Surtout, le passe est d'application immédiate et n'exclut pas, le cas échéant, la première solution. Si l'on se rallie à cette stratégie, ce qui est mon cas, il reste à en préciser les contours. Les rédacteurs du texte initial, pensant sans doute que, pour parler fort, il faut avoir un gros bâton, ont eu la main lourde. Le Conseil d'État a déjà freiné quelques ardeurs sur le montant des amendes ou le droit du travail. Nous devons apporter notre pierre à l'édifice et, en tant qu'élus proches du terrain, faire en sorte que le passe sanitaire ne soit pas la première étape de notre plan de relance industrielle, la relance de la production de paperasserie.

La vaccination pour tous, c'est la liberté pour tous. Les droits de chacun doivent être respectés, les contraintes excessives évitées, mais à condition de ne pas mettre en danger la santé d'autrui et de ne pas oublier que le corollaire de la liberté, c'est la responsabilité.

Et si j'ai également toujours déploré votre méthode de gouvernance, je ne me suis jamais opposé à vos choix en matière de lutte contre la covid-19. J'aurais espéré qu'après un an et demi de pandémie

Alors que la France est en retard par rapport à ses voisins en matière de vaccination, alors que les doses manquent encore pour vacciner les quelque 20 millions de Françaises et de Français qui ne le sont pas, alors que le Gouvernement fait, mois après mois, la démonstration de son manque d'anticipation, le Président de la République continue de décider seul de mesures qui menacent gravement les libertés publiques. Madame la ministre, nous sommes fatigués de cette morgue, de ce paternalisme, de cette arrogance. En vous adressant aux Français comme à des enfants, en n'admettant jamais vos nombreuses erreurs, en multipliant les propos à l'emporte-pièce sur les masques, les vaccins, le passe sanitaire, vous dépréciez- hélas ! -méthodiquement la valeur de la parole publique. La défiance qui s'accroît depuis les premiers jours du quinquennat atteint un niveau invraisemblable. Comment convaincre des citoyens chauffés à blanc de la nécessité de se faire vacciner ? Ils sont tellement exaspérés qu'ils tombent dans les bras des populistes et des complotistes les plus abjects, qui usent de comparaisons à vomir et accentuent les fractures de la société. Ce cercle vicieux, vous n'avez malheureusement pas fait grand-chose pour le rompre, loin de là. Votre passe sanitaire, inapplicable, montera les gens les uns contre les autres.

Que prévoyez-vous pour rapprocher les plus jeunes de la vaccination ? Et surtout, quelles mesures allez-vous prendre pour enfin déployer la vaccination dans les quartiers populaires ? Les inégalités sociales face au vaccin sont criantes. C'est l'ignorance autant que la défiance qu'il faut combattre.

Vous ne laissez même pas la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de se faire vacciner à temps. Vous instaurez le contrôle de tous par tout le monde, selon un dispositif juridiquement bancal, et ce malgré les alertes du Conseil d'État et de la Défenseure des droits. Vous imposez des amendes délirantes, équivalentes à celles qui sont applicables en cas d'usurpation d'identité, par exemple. Dans le même temps, faisant fi des recommandations sanitaires, vous autorisez l'abandon du masque dans les lieux soumis au passe sanitaire.

Vous n'écoutez aucun représentant des oppositions, alors même que celles-ci sont toutes d'accord contre vous. Vous ne consultez pas ou vous faites semblant ; vous n'associez que très peu les collectivités locales. Contrairement à ce que vous semblez croire, tout cela ne nous fait pas gagner en efficacité, très loin de là, hélas ! Bien des régimes parlementaires, à commencer par l'Allemagne, enregistrent de meilleurs résultats que nous dans la gestion de l'épidémie sans s'asseoir pour autant sur la délibération démocratique. Alors, madame la ministre, j'espère que vous retiendrez au moins les apports de bon sens du Sénat. Je pense en particulier aux mesures d'isolement. Pour les écologistes, en l'état, cela reste insuffisant. Le texte permettrait trop d'atteintes aux libertés publiques. Il découle de trop de promesses bafouées et créerait trop de divisions. Nous appelons le Gouvernement à « mettre le paquet » sur la stratégie vaccinale plutôt que de contraindre trop brutalement et de diviser. Nous appelons enfin à lever les brevets sur les vaccins et à favoriser leur diffusion mondiale. Tous les efforts que nous faisons, toutes les restrictions que nous nous imposons devront se poursuivre tant que nous permettrons au virus de circuler largement dans le monde, tant qu'il mutera et que des variants apparus aux quatre coins du monde, résistant à nos vaccins, reviendront frapper à notre porte. L'égoïsme vaccinal des pays occidentaux, les gestions nationales de l'épidémie de covid-19 sont des impasses sanitaires. Il est grand temps de sortir du cadre national pour enrayer, enfin, la pandémie.

compris le contrôle en référé quasi instantané du tribunal administratif- il n'y a donc pas du tout de déni de justice. De par la rapidité d'application et le caractère direct

qui en font une solution immédiate, il nous reste probablement une bonne quinzaine de millions d'injections à réaliser pour arriver à un taux de couverture suffisant, en tenant compte des personnes qui n'ont pas encore reçu leur première dose et de celles qui ont reçu la première, mais doivent attendre la seconde. Instaurer

Nous avons un espoir. Nous avons cette chance inouïe de disposer de plusieurs millions de doses proposées gratuitement à la population- faut-il le rappeler ? - pendant que, comme l'indiquait mon collègue Bernard Fialaire, dans de nombreux pays n'ayant pas atteint notre degré de développement, nombreux sont ceux qui les réclament ou qui meurent de ne pas les avoir reçus. Je pense bien sûr aux Tunisiens, qui connaissent des heures sombres et à qui nous exprimons toute notre amitié et notre solidarité. Pendant qu'ils comptent leurs morts, faute de bouteilles d'oxygène et de vaccins en nombre suffisant, nous en sommes toujours à débattre de l'efficacité et de la sécurité de la vaccination. Bien sûr, il faut écouter ceux qui doutent, les sceptiques, les réticents. Il faut dialoguer avec eux, faire preuve de pédagogie, leur redire que toutes les phases de test et les procédures d'autorisation sont respectées, que la pharmacovigilance assure une surveillance continuelle des éventuels effets secondaires. Le soin, malgré tout, reste basé sur la confiance et la médecine sur des faits scientifiques, que l'on ne peut balayer sur la base de supputations sans fondements. Mais il faut aussi être intraitable vis-à-vis des plus virulents, ceux qui dégradent les centres de vaccination, qui menacent les personnes y travaillant, qui comparent notre pays à une dictature et notre système de santé à la Shoah.

Personne n'a l'obligation de tout maîtriser ou de tout comprendre. En revanche, chacun a l'obligation éthique et morale de se forger un avis à partir des faits. De ce point de vue, la vaccination nous protège contre les formes graves du virus et en limite la circulation, comme l'absence quasi totale de patients vaccinés en réanimation en témoigne. L'immunité collective est un objectif vers lequel nous devons tendre et les mesures de ce texte y contribuent. Face à l'arrivée du variant delta, dont la charge virale est multipliée par mille et dont le taux de contamination est de 60 % plus élevé que celui du virus malheureusement et de toute urgence prendre de nouvelles mesures si nous voulons contenir une quatrième vague, qui risque de nous submerger et de nous obliger au confinement, ce que personne ne souhaite. Cette pandémie, par sa violence et son extraordinaire résistance, nous impose des ajustements perpétuels. Les nouvelles mesures de ce texte en choquent certains, vu le nombre de messages que nous recevons dans nos boîtes mail, car elles contraignent l'accès aux activités du quotidien. Il est vrai que ces ajustements touchent à certaines de nos libertés

Si l'on veut un statut vaccinal complet au 15 septembre prochain, il faudrait avoir reçu sa première dose avant le 18 août. Or certains centres ne proposent pas de créneaux avant la fin du mois d'août. À ce sujet, madame la ministre, il conviendrait de confirmer que les personnes soumises à l'obligation vaccinale auront un accès prioritaire au vaccin, afin de pouvoir se mettre en règle au plus vite. Nous devons privilégier l'incitation et récompenser ceux qui sont engagés dans la démarche de la vaccination. Quand on sait que l'immunité acquise est forte dès trois semaines après la première injection, une tolérance ne pourrait-elle pas être accordée aux primo-vaccinés ?

le taux de vaccination de la population et des soignants demeure insuffisant- c'est une réalité. L'obligation vaccinale n'est pas une stigmatisation, comme on l'entend souvent. Elle existe déjà contre l'hépatite B et évolue en fonction de la situation sanitaire. Elle vise à protéger les soignants, mais aussi à répondre, comme le disait notre rapporteur pour avis, à leur « exigence d'exemplarité » et à leur « devoir éthique » vis-à-vis des personnes vulnérables qu'ils s'engagent à protéger au quotidien. Je suis donc favorable à l'obligation vaccinale, et proposerai même de l'étendre à d'autres professions. Je m'interroge par ailleurs sur les conditions de contrôle du passe sanitaire dans les restaurants et les cafés. Je serai favorable à ce que la responsabilité porte sur le consommateur, plutôt que sur l'exploitant, et que les contrôles soient effectués par des personnes habilitées à le faire. Enfin, je ne peux terminer mon propos sans évoquer le délai si court qui nous est octroyé pour l'examen de mesures d'une telle importance. Si nos marges de manoeuvre sont comme souvent limitées, nous aurions tout de même apprécié de pouvoir prendre le temps de la réflexion et du débat. Toutefois, vous l'aurez compris, madame la ministre, je partage la philosophie du texte et la nécessité de ces mesures de freinage de la circulation virale et de déploiement massif de la vaccination.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, d'emblée, je souhaite vivement contester la précipitation de ce débat. Celle-ci ne permet pas d'examiner sérieusement les dispositions proposées, qui ont d'ailleurs évolué au fil des jours.

Je ne sais comment nous devons interpréter ce départ précipité du ministre, qui n'a même pas pris le temps d'écouter la discussion générale, en particulier les interventions des groupes.

La démocratie, le pluralisme, c'est savoir écouter, prendre en compte et parfois concéder et reconnaître ses erreurs. Oui, nous savons que le variant delta se répand vite, et ce depuis de nombreuses semaines. Oui, nous savons qu'en France les contaminations repartent vivement à la hausse. Nous savons aussi que la vaccination est le rempart efficace pour éviter les hospitalisations et les réanimations. réanimations. C'est un outil formidable pour venir à bout de l'épidémie. À ce titre, nous demandons que le vaccin soit reconnu comme grande cause nationale et mondiale et, donc, que les brevets soient levés. Mais il faut des moyens pour aller au plus près de la population non vaccinée, souvent par abandon social ou manque d'information. Informer, convaincre, mobiliser tous les acteurs de la société, telle est la clé d'une vaccination pour tous. C'était, peu ou prou, la position de M. Olivier Véran. Alors, pourquoi un tel revirement ? Comment ne pas être surpris par cette volonté soudaine de culpabiliser notre peuple, de le diviser, de le fracturer ? C'est M. Olivier Véran, lui-même, qui a refusé les vaccinodromes en janvier dernier. C'est lui qui a fait le choix d'une vaccination progressive de la population, rappelant durant des semaines que les jeunes ne risquaient pas tant et pouvaient attendre. Qui a fait le choix de commander massivement le vaccin AstraZeneca, qui fut sévèrement critiqué jusqu'à être interdit dans plusieurs pays ? La campagne vaccinale fut même suspendue en France. En mai et en juin dernier, la vaccination a décollé et la suspicion a reculé.

De plus, pourquoi produire un argumentaire culpabilisateur à outrance, alors que les doses ne sont pas disponibles pour parvenir rapidement à l'immunité collective ? Madame la ministre, l'analyse que nous développerons au cours des débats est la ce projet de loi et le discours d'Emmanuel Macron sont un aveu d'échec manifeste. Notre peuple n'est pas assez vacciné, non pas parce qu'il est récalcitrant, mais parce que vous n'avez pas mis en oeuvre les moyens nécessaires. Ensuite, et « en même temps », le Président de la République utilise ce moment pour accentuer la dérive autoritaire de son pouvoir et placer notre pays sous une cloche libérale. Le 12 juillet dernier, il a mêlé sa nouvelle réponse sécuritaire pour contrer la crise sanitaire à la confirmation ou à l'annonce de coups de force antisociaux. Dans son intervention, l'autoritarisme apparaît comme le point commun des différents aspects de la politique du pouvoir actuel. La prolongation de l'état d'urgence sanitaire du 30 septembre au 31 décembre 2021 symbolise le maintien d'un état d'exception. L'instauration du passe sanitaire est un outil de division de notre peuple. Le respect du droit et de l'égalité est à préserver. Comme d'innombrables juristes, associations et syndicats, s'est vivement inquiétée et a énoncé dix recommandations précises, importantes pour préserver les libertés et le droit face à vos propositions. J'aimerais connaître votre réponse détaillée à ces interpellations. Le passe sanitaire est, selon nous, vicié dès le départ. Qui dit passe sanitaire dit contrôle d'identité ... Madame la ministre, soit vous faites contrôler l'identité des gens par des personnes non assermentées et c'est une dérive inacceptable, soit vous permettez d'intensifier les contrôles de police inopinés dans les restaurants, dans les cinémas, dans les salles de sport, dans les transports, ou encore à domicile dans le cadre des procédures d'isolement. Est-ce là le modèle de société que vous portez ? Une société de suspicion, de contrôle permanent !

Mais pourquoi brandir, là aussi, la menace de la suspension et du licenciement ? L'obligation d'isolement soulève également d'importants problèmes de droit. Nous refusons qu'une mesure privative de libertés- car c'est de cela dont il s'agit -puisse découler d'un seul test positif, sans décision de justice. Par ailleurs, comment ne pas constater une nouvelle fois la discrimination à l'égard des moins favorisés, qui ne peuvent respecter l'isolement du fait de conditions de logement précaires ? Enfin, madame la ministre, comment ne pas s'alarmer du changement de donne concernant le système d'information national de ? Réservé au personnel de santé, il sera consultable, demain, par toutes les catégories de personnes habilitées à effectuer des contrôles. La préservation des données personnelles et le secret médical sont foulés aux pieds par votre projet. Madame la ministre, nous voterons contre ce texte, même provisoirement assoupli par le Sénat. Sous le couvert d'un combat pour la vaccination, il accélère en effet le développement d'un projet de société attentatoire aux libertés et aux droits des salariés, sans armer notre pays face aux pandémies.

mes chers collègues, les sénateurs centristes abordent le débat sur la réponse à la crise sanitaire en suivant deux lignes directrices.

Ils refusent d'alimenter une passion française pour le droit pénal et de brandir la menace du licenciement, là où la suspension du contrat de travail et des salaires nous semble déjà très suffisante. Quelques mots sur notre diagnostic : la crise de la covid-19 dure depuis dix-huit mois, la maladie est installée probablement pour longtemps et le virus ne connaît pas les frontières. Nous avons demandé, hier matin, au professeur Jean-François Delfraissy de nous aider à nous projeter sur le long terme. Il nous a exprimé les doutes et les incertitudes de la communauté scientifique, et nous a présenté les deux thèses privilégiées. Pour les optimistes, après une vaccination généralisée, le virus continuera d'évoluer- avec peut-être une ou deux mutations encore -tout en perdant progressivement sa capacité à contaminer ou, plus simplement, sa dangerosité.

La réponse nécessite de choisir entre de mauvaises ou de très mauvaises solutions. Nous abordons cette question avec humilité, en étant conscients que nous sommes dans une société, sinon de peur, au moins de défiance, où l'émotion l'emporte régulièrement sur la rationalité et où l'individualisme a souvent, vous le savez bien, pris le pas sur le collectif. Cela nous conduit à ne pas trop asséner de vérités, à exprimer des réponses mesurées, dont nous devons admettre qu'elles pourront évoluer, à cultiver en définitive une éthique du doute et du respect des opinions.

Tenons aussi compte du fait que nous sommes dans une société où chaque vie est essentielle. Il n'est pas possible de raisonner sur une forme d'acceptation d'un nombre de morts ou de malades graves, même s'il n'est interdit à aucun d'entre

La vaccination obligatoire générale a le mérite de répondre clairement à l'enjeu de santé publique. Le dispositif est simple, précis, conforme à une autre passion française, celle de l'égalité. Il est aussi pédagogique.

possible ? Nos concitoyens accepteront-ils une telle mesure ? Comment l'État la fera-t-il respecter ? Si la vaccination devenait obligatoire, l'État engagerait évidemment sa crédibilité sur l'exécution de ces dispositions.

La proposition de rendre obligatoire la vaccination des soignants ne fait aucune difficulté dans notre groupe. Il s'agit, à nos yeux, de la simple application de règles éthiques. C'est aussi une question de confiance dans notre pacte social. Reste la question du passe sanitaire

À l'Assemblée nationale, le passe sanitaire a été décrit comme un outil de liberté, une incitation à se faire vacciner, pour permettre à chacun d'entre nous d'avoir une vie normale. vue psychologique, les prises de rendez-vous massives en vue de la vaccination, dans les heures qui ont suivi l'intervention du Président de la République, l'ont démontré. Je voudrais cependant attirer votre attention, mes chers collègues, sur la limite de cet exercice, en tout cas la contradiction ou l'ambiguïté du passe sanitaire nous est proposé à titre incitatif, pour favoriser la vaccination, alors que sa vocation devrait être sanitaire. Le passe sanitaire n'est pas, à l'inverse de la vaccination, une réponse de santé publique en tant que telle. Il ne soigne pas.

des affaires sociales, mené par les rapporteurs Philippe Bas et Chantal Deseyne. J'insiste sur le changement de logiciel. En décidant, si le texte est voté,

Madame la ministre, l'examen du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire se déroule dans un agenda excessivement contraint, signe d'un manque d'anticipation de votre part, qui donne une impression de chaos, au moment où nous avons tous collectivement besoin d'un cap clair. Nous sommes convaincus, au sein du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat, que vous en viendrez nécessairement à la position qui est la nôtre ; pour nous, le seul chemin aujourd'hui envisageable pour prendre la main sur l'épidémie est celui d'une vaccination universelle. Nous faisons ce choix pour que chacun puisse être protégé et protège les siens, tout en jouissant de ses droits fondamentaux. Plusieurs institutions du champ scientifique et médical se sont d'ores et déjà prononcées en faveur de l'obligation vaccinale généralisée. C'est notamment le cas de l'Académie nationale de médecine, qui a pris position dans un communiqué, le 19 juillet dernier, jour de présentation en conseil des ministres du présent projet de loi. Je vous rappelle d'ailleurs qu'elle s'était prononcée publiquement en faveur du port du masque dès avril 2020, quand le Gouvernement soutenait encore qu'il ne servait à rien en population générale. Nous espérons que l'alignement du Gouvernement sur ces positions n'interviendra pas trop tard. En attendant, nous voilà contraints de travailler sur une politique qui menace d'être inopérante, incohérente et liberticide. Et c'est si flagrant que vous vous retrouvez dans la position de devoir procéder à ajustement sur ajustement, dans l'espoir de consolider un édifice de plus en plus bancal. C'est tout particulièrement le cas pour les modalités relatives à l'instauration d'un passe sanitaire, qui aboutissent à la stigmatisation des professionnels intervenant dans le secteur de la santé. Vous créez une nouvelle obligation vaccinale, mais seulement pour certaines catégories professionnelles, avec un système de sanctions parfois très lourdes,

La définition du périmètre de votre dispositif est particulièrement large ; les critères sont flous, à la limite d'un certain arbitraire. Sont visées par l'obligation que vous entendez mettre en place des catégories de personnes définies non seulement par leur profession, mais aussi par leur lieu d'exercice professionnel. Vous dressez une sorte d'inventaire à la Prévert, allant des aides à domicile aux sapeurs-pompiers, en passant par les élèves et les psychanalystes. En revanche, policiers et professeurs ne sont pas concernés par l'obligation vaccinale, alors même que ces derniers travaillent tout particulièrement au contact de publics au sein desquels la circulation du virus est forte et incontrôlée. Signe du caractère hasardeux de votre démarche, vous prenez le risque de fracturer la société française en désignant des professionnels qui pourraient en plus faire l'objet d'un traitement différencié, évoluant au gré des rectifications que vous y apporterez. Le Gouvernement a en effet introduit une nouvelle disposition annoncée la veille par la ministre du travail : la possibilité pour le salarié de convenir avec son employeur de prendre des réductions de temps de travail (RTT) ou des jours de congés pour éviter une suspension du contrat de travail. C'est dire si la mesure initiale était pertinente ! Vous vous donnez beaucoup de mal, et vous nous donnez beaucoup de mal, pour imposer sans le dire une vaccination généralisée. Dans cette pandémie qui n'en finit pas, le courage politique consisterait à dire à tous les Français qu'ils doivent obligatoirement se faire vacciner, quel que soit leur environnement professionnel. Le courage politique serait d'affirmer que se faire vacciner pose un acte de solidarité, de fraternité même, en ce qu'il induit l'intérêt de l'autre au-delà de l'intérêt propre à chacun et en ce qu'il positionne l'individu non pas comme une pièce unique et autocentrée, mais comme un citoyen conscient du rôle qu'il doit jouer dans un moment crucial pour le groupe auquel il appartient. Le courage politique serait d'assumer une décision de vaccination universelle obligatoire, qui permettrait d'assurer la concorde au sein de la société française. Ce ne sont pas les libertés publiques que l'on doit combattre : la liberté de circulation et d'accès aux biens et aux services, l'égalité de traitement et la protection contre l'arbitraire ne sont pas la maladie ! Nous ne voulons pas d'un passe liberticide. Ce que nous souhaitons, c'est atteindre l'immunité collective- celle-ci est fixée à un taux de population vaccinée contre la covid-19 de 90 %, du fait des variants en circulation, tout particulièrement le variant delta. Nous nous inscrivons également dans une démarche de santé publique claire, assise sur des connaissances médicales et scientifiques.

C'est d'une politique de santé publique dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous attendons des mesures et des textes pertinents, de même que les moyens humains et budgétaires nécessaires pour lutter contre cette maladie et assurer la protection sociale dans une démarche de lutte contre les inégalités territoriales et sociales, pour assumer son devoir d'aller vers les publics les plus éloignés de la vaccination. Sans moyens supplémentaires, les mesures envisagées s'avéreront encore plus dures pour les publics précaires. Or nous savons que ce sont eux qui ont le moins accès aux vaccins. Nous sommes confrontés à un problème de santé qui remet fondamentalement en cause l'équilibre de la société. Le pays est prêt à des efforts, fussent-ils coûteux- il l'a démontré depuis plus d'un an. Poursuivre l'objectif de vaccination obligatoire universelle sans l'assumer, c'est autre chose : c'est le pire des choix Vous avancez masqués avec l'outil pervers du passe sanitaire, imposant tout en la dissimulant, une obligation vaccinale généralisée. Le caractère trouble de votre démarche est perçu par la population il suscite un rejet qui met en péril non seulement l'efficacité de la politique de lutte contre la covid-19, mais aussi les assises de notre système politique tout entier. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de solidarité et d'unité. Et cela passe nécessairement par la vaccination généralisée

il faut se rendre à l'évidence : nous n'en avons pas terminé avec cette pandémie. La stratégie de vaccination est essentielle, mais elle n'est pas unique.

la devons à tous les Français, non pas seulement à ceux qui comprennent la nécessité de la vaccination, mais aussi à ceux qui peuvent avoir des réticences. Nous devons relayer leurs interrogations car, même si nous ne les comprenons pas toujours, elles peuvent être légitimes. En tout cas, nous devons leur répondre autrement que par des injures ou par des invectives. Pour respecter cet

voilà une dizaine de jours, à annoncer que nous saisirions le Conseil constitutionnel, non pas pour dresser un nouvel obstacle sur le chemin de ce texte, mais tout simplement pour indiquer aux Français que nous allions prendre toutes les précautions, toutes les garanties

chacun ici, ce soir, a rappelé la gravité de la crise sanitaire que nous vivons. Les chiffres ont été égrainés, nous les avons à l'esprit. Mais, depuis dix-huit mois, nous nous retrouvons ici régulièrement. madame la ministre, dans la gestion de cette crise, a commis une triple faute. La première, c'est l'infantilisation, a considéré que les Français devaient être traités comme des enfants. Ce furent les attestations pour avoir le droit de sortir ; ce sont désormais, au fil du temps, chaque fois, des leçons qui sont assénées, comme si chacun ne pouvait pas entendre la gravité de la situation.

que même ses propres ministres, ses équipes ne savaient pas précisément ce qui allait être annoncé, l'intendance suivant. De fait, les mesures annoncées étaient évolutives, puisqu'elles ne pouvaient pas trouver leur application. faute : les errements et les revirements. C'est peut-être ce qui est le plus gênant, car, aujourd'hui, la confiance dans votre parole a singulièrement fondu. fondu. À cette même tribune, il nous a été tenu des propos définitifs sur le passe sanitaire, qui ne serait jamais appliqué pour des actes de la vie quotidienne, mais aussi, au gré des étapes et sans vouloir rappeler de cruels souvenirs, sur l'inutilité de porter des masques. Au fil du temps, chaque fois, la parole publique a été dévalorisée. Tout cela a conduit à un triple désastre un désastre sanitaire, un désastre démocratique et un désastre social. Un désastre sanitaire, d'abord. Nous le constatons : les contaminations repartent,

les propos d'une autorité constitutionnelle, la Défenseure des droits, qui souligne notamment l'inintelligibilité des règles. Car, si demain un Français est capable d'expliquer ce qu'il est possible de faire ou pas, nous pourrons alors le saluer.

une forme de discrimination à l'emploi entre les vaccinés et les non-vaccinés, ce qui aura évidemment pour effet de mettre en grande difficulté les catégories sociales les plus défavorisées, celles-là même dont nous savons qu'elles sont les moins vaccinées.

tout en indiquant qu'elle serait l'étape suivante. Mais pourquoi attendre l'étape suivante, puisque nous savons qu'il faut du temps pour la mettre en place ? Nous proposons un certain nombre de mesures qui pourront être effectives dès demain, sanctionnables

devant le Parlement. Sauf que nous aurons, encore une fois, pris du retard et, encore une fois, manqué l'occasion de permettre à nos concitoyens de sortir de cette crise.